Si les éléments parcellaires qui nous ont été transmis à ce stade laissent à penser que le Gouvernement a bien l'intention de respecter la trajectoire fixée par la loi d'orientation des mobilités (LOM), avec 2,782 milliards d'euros de dépenses- nous y reviendrons dès vendredi en deuxième partie il paraît déjà clair que les recettes prévues pour financer ces dépenses ne sont pas crédibles, compte tenu de la poursuite de la crise sanitaire. C'est en particulier le cas des 230 millions d'euros d'écocontribution du transport aérien et des 278 millions d'euros de produit des amendes radar. C'est pourquoi les rapporteurs spéciaux pour les crédits des transports terrestres de la commission des finances proposent au Sénat d'adopter un amendement visant à relever

La TICPE est en effet une recette fiable sur laquelle l'agence pourra à coup sûr compter. Si la situation sanitaire s'améliore fortement et que les autres recettes de l'Afitf

Monsieur le ministre,

du montant maximum de prélèvement des redevances. Ce dispositif limite la capacité d'action des agences, alors même que le onzième programme élargit leur champ d'action et que la crise du covid-19 nécessitera non seulement un accompagnement supplémentaire des collectivités

a été estimé à environ 2 millions d'euros par an lors des assises de l'eau. Cet amendement vise à supprimer le plafond mordant des agences de l'eau afin de mettre ces dernières en mesure de faire face aux nombreux défis présents et à venir tels que l'adaptation au changement climatique, l'appui à la transition agricole, la surveillance de la qualité physico-chimique des eaux ou encore les subventions aux travaux d'assainissement non collectifs non encore réalisés. Au-delà des mesures de court terme, il est particulièrement nécessaire que les agences de l'eau puissent oeuvrer efficacement à la résilience du secteur face aux crises actuelles et futures à travers l'entretien et le renouvellement du patrimoine, l'adaptation au changement climatique, laquelle nécessitera des travaux d'interconnexion pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable, la réutilisation des eaux non conventionnelles et

et la modernisation des stations d'assainissement et 30 millions d'euros pour l'hygiénisation des boues. Il s'agit d'améliorer la résilience de l'alimentation en eau potable, notamment face aux risques de sécheresse,

Constatant une diminution des ressources pour Action Logement, le Gouvernement a créé une taxe supplémentaire sur les contrats d'assurance et lui en a affecté le produit. Or, deux ans plus tard, l'État revient sur sa parole et nous propose ici de supprimer cette compensation.

Action Logement est, avec ses partenaires, un acteur clé pour appréhender la période de relance, alors que la crise sanitaire que nous traversons accentue les difficultés d'accès au logement et

Il y a vraiment des choix à faire : Action Logement ne peut pas être la boîte à outils à tout faire du Gouvernement en matière de logement, jusqu'à financer les aides personnalisées au logement.

faire à Action Logement avec la PEEC n'est peut-être pas non plus une bonne politique

les reports massifs des parieurs constatés sur les championnats de football maintenus dans le reste du monde et le maintien de toutes les compétitions sportives à huis clos lors de la seconde vague ont permis de préserver l'activité des entreprises de jeu.

est fortement menacé par l'hypothétique renégociation des contrats entre diffuseurs, depuis les annonces du groupe Mediapro sur le championnat professionnel de football français.

sur les sommes misées sur les paris sportifs. En effet, le plafond actuel de la taxe sur les paris sportifs ne représente que 31 % des recettes fiscales prévues en 2021. Ce rehaussement offrira donc une visibilité accrue à l'Agence nationale du sport pour assurer la solidarité financière directe entre le sport professionnel, le sport amateur et le sport pour tous.

Elle a rappelé qu'il était trop tôt pour évaluer les conséquences du conflit avec Mediapro, mais nous a assurés que l'Agence nationale du sport percevrait bien les ressources annoncées, même en cas de renégociation du contrat.

aux acteurs du monde sportif la mise en place d'un dispositif Pass'Sport en 2021, géré par l'Agence nationale du sport et financé par l'État à hauteur de 100 millions d'euros.

de soutenir les fédérations sportives et les clubs, alors que ceux-ci font face à une crise sans précédent : les chiffres les plus récents font apparaître des pertes supérieures à 350 millions d'euros.

Le Président de la République a donc annoncé une enveloppe de 100 millions d'euros pour compenser les pertes de billetterie, mais, encore une fois, rien n'est inscrit au budget 2021.

honorer ses échéances. Il n'est donc pas abusif, malgré les engagements oraux du Président de la République, de craindre de se retrouver dans la même situation qu'au milieu des années 2000, avec la défaillance de MP & Silva. Dans ce climat défavorable, nous avons, comme d'autres groupes ou collègues, décidé de proposer cette mesure, parce que la manne de Mediapro, estimée à près de 40 millions d'euros de taxe Buffet par an, est devenue largement hypothétique.

de Ligue 2 : on peut assister, d'ici à la fin de la saison sportive, à des dépôts de bilan de clubs, avec tous les dégâts médiatiques que cela pourrait provoquer.

Or cette baisse de plafond des ressources est incohérente avec l'ambition affichée par le plan de relance et compromet sa mise en oeuvre dans les territoires, au plus près des entreprises. En ces temps de crise sanitaire, sociale et économique, les CCI ont plus que jamais un rôle d'accompagnement à jouer auprès des TPE et des PME. Il s'agit donc de supprimer l'alinéa 13 afin de préserver le maillage territorial des CCI.

le plafonnement, mais sans prévoir de prélèvement sur les réserves de l'INPI.

Le premier argument s'opposant à la mise en application de la loi est que la recette susvisée est inscrite à l'article du code de l'environnement auquel s'applique le plafonnement précisé à l'article 46 de la loi de finances pour 2012. Or cette recette ne constitue pas une redevance en tant que telle ; seul son calcul est basé sur une redevance existante.

l'avis du Gouvernement ? La mise en plafond de la possibilité de majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau reviendrait à remettre en cause l'effectivité du plafond des taxes affectées aux agences de l'eau. Or nous considérons que le dispositif de plafonnement global des redevances offre déjà de la souplesse aux agences, car il est adapté à leur situation : ce sont les seuls organismes disposant d'un système de plafonnement individuel couplé à un système de péréquation, ce qui permet de garantir le niveau de recettes et de moduler le taux de redevance en fonction des caractéristiques du bassin.

présenter l'amendement n° I-325 rectifié. Cet amendement vise à compenser, pour le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), les moindres recettes perçues en 2019 en raison de l'exonération de taxe pour frais de CMA dont ont bénéficié les entreprises ayant réalisé moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Le plafond de recettes affectées allouées aux CMA, fixé à 203,1 millions d'euros, est en effet décliné en plafonds régionaux : selon le dynamisme de la base fiscale, certaines régions perçoivent une recette inférieure au plafond, sans que d'éventuels trop-perçus par d'autres régions puissent leur être transférés ponctuellement, puisque ces derniers sont versés au budget général. La perte de recettes pour le réseau s'élève au total à 2,7 millions d'euros. Il est proposé de compenser cette perte par un relèvement temporaire, pour un an, du plafond de taxes affectées de 2,7 millions d'euros. Il s'agit d'une mesure d'équité, mais également d'efficacité, le réseau des CMA étant fortement mobilisé depuis le début de la crise pour accompagner les artisans. Aides à la numérisation, communication sur les aides, soutien psychologique, dizaines de milliers d'appels passés sont autant d'actions largement reconnues par les acteurs de terrain et menées avec des moyens constants, voire en baisse dans certaines régions. Cet amendement vise donc à corriger un effet de bord de l'exonération pour les petites entreprises en permettant au réseau de percevoir l'intégralité de la taxe affectée prévue par la loi.

soit 2,7 millions de moins que le plafond général, et ce malgré un rendement de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat (TFCMA) de 209,4 millions d'euros en 2019. Cette « perte » n'est en rien imputable aux chambres de métiers et de l'artisanat elles-mêmes : elle est le résultat de l'exonération de TFCMA voulue par le Gouvernement pour les entreprises ayant réalisé moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires.

de ressources. C'est pourquoi cet amendement vise à relever le plafond de 2,7 millions d'euros pour 2021 afin de compenser cette même somme manquante dans le versement

national du plan Écophyto à hauteur de 41 millions d'euros, afin de viser l'objectif de réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici à 2025. Engagé en 2018, le plan Écophyto a permis de mettre en place de nombreuses actions structurantes, telles que le réseau Dephy, les fermes pilotes, le bulletin de santé végétale et de nombreux autres projets de recherche et d'innovation. Ce plan a été élargi à 2015, puis consolidé en 2018 pour devenir Écophyto II+. Les exigences sociétales en matière de sécurité alimentaire sont croissantes. à tous, dite Égalim, prévoit de nombreux dispositifs visant à améliorer les conditions sanitaires et environnementales de production. Il ne faut donc pas relâcher les efforts. Dans cette perspective, le budget doit prévoir les moyens suffisants pour accompagner les agriculteurs

créée et mise en oeuvre au titre de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, il est important que les bénéfices de la valorisation du sport professionnel français puissent intégralement bénéficier au sport amateur, ce qui alimentera un cercle vertueux pour le sport français. Je précise que l'adoption

Au regard de ces annonces, de la situation économique catastrophique dans laquelle se trouvent les clubs de sport professionnels masculins et féminins- plus de billetterie, des partenariats qui revoient leur participation à la baisse, des collectivités en difficulté -et de la situation d'urgence que nous affrontons, il me semble que les conditions sont pleinement réunies pour qu'un groupe de travail soit constitué dans les plus brefs délais et qu'une solution soit trouvée d'ici à la fin de l'examen du projet de loi de finances pour 2021

Cet amendement vise à simplifier le processus d'établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l'assurance au pouvoir de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

perçoit des recettes dont le montant fluctue en fonction de l'activité économique, en particulier la taxe d'aménagement du territoire, qui est assise sur le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier concédé, les amendes radar et l'écocontribution sur les billets d'avion. Il en résulte, chaque année, une imprévisibilité quant aux recettes réelles qui seront perçues par l'Afitf, alors même que celle-ci est engagée dans le financement de travaux d'infrastructures sur le temps long. En raison de la crise sanitaire actuelle, les pertes de recettes pour l'Afitf au titre de l'année 2020 sont évaluées à 500 millions d'euros et font l'objet d'une compensation partielle dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative et du quatrième projet de loi de finances rectificative. Pour 2021, les prévisions de recettes sur lesquelles le budget de l'Afitf est construit paraissent sujettes à caution en raison de la poursuite probable des impacts de la crise sanitaire sur le trafic routier et aérien. L'affectation des taxes sur les autoroutes et l'aérien et des amendes radar à l'Afitf a une vertu pédagogique, en

tout en faisant de la part de TICPE versée à l'Afitf une variable d'ajustement, dont le montant sera modulé en fonction de celui des autres recettes perçues, en vue d'équilibrer le budget

face aux risques naturels. Enfin, il améliore la connaissance du risque par des études et des campagnes d'information. Il est principalement alimenté par une part des primes pour la couverture du risque de catastrophe naturelle qui figurent dans les contrats d'assurance. Compte tenu de la multiplication des aléas climatiques, ce fonds revêt une importance stratégique majeure, comme l'atteste son usage au moment de diverses catastrophes naturelles en outre-mer

indiquait que le fonds Barnier était « la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels, menant une véritable politique incitative pertinente au profit d'une meilleure couverture des

Que fera-t-on des 600 millions d'euros de trésorerie du fonds s'il est intégré au budget de l'État ? Que deviendront les crédits déjà délégués aux départements pour verser les subventions sur lesquels l'État s'est engagé et qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros ?

sur le modèle du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques (Cipac). Cela permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu les dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement, dans le but d'améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

présenter l'amendement n° I-630 rectifié . Les cafés, hôtels, restaurants, discothèques (CHRD) et les entreprises du tourisme sont dans une situation économique d'une gravité extrême, compte tenu de l'obligation de fermeture administrative et de l'interruption brutale des flux touristiques. Cette situation s'est encore accentuée avec le deuxième confinement.

puissent bénéficier à titre exceptionnel d'une réduction de 50 % du montant de leur contribution à l'audiovisuel public.

et Territoires s'oppose à la fragilisation continue du service public de l'audiovisuel, qui s'est traduite par la suppression de plus de 2 000 postes à France Télévisions depuis 2012, la disparition de France Ô, qui constitue une véritable perte culturelle et qui va, par ailleurs, à rebours des engagements du Président de la République.

je crois qu'un audiovisuel public fort, qui fonde la mise en oeuvre de ses programmes sur la raison, la science et la diversité des points de vue, dans le respect des règles de la République, serait